départements. Comment ne pas leur donner raison ? La Guyane et la Martinique avaient été consultées, tout comme nos concitoyens alsaciens, qui avaient d'ailleurs rejeté le projet de collectivité unique.